Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et au respect du temps de parole. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour le groupe Les Républicains.

doit maintenant faire face. Nous étions réunis hier, en Avignon, pour rendre un dernier hommage au commandant Éric Masson, un « homme de bien », comme vous l'avez justement dit. Hommage lui soit encore rendu ainsi qu'à toutes les forces de l'ordre de notre pays, qu'il faudrait enfin apprendre à aimer ! La République a fait corps autour de ce crime de trop, et je pense que tout un département vous en remercie. Cependant, nos concitoyens ne supportent plus ce goutte-à-goutte de criminalité qui diffuse maintenant jusque dans nos campagnes. Bédarrides, où vivait Éric Masson, Cavaillon, ma ville, où a eu lieu il y a quelques jours un règlement de compte similaire, les petites villes et les villages qui représentent une Provence heureuse ne veulent pas devenir la base arrière de Marseille. n'acceptent pas cette nouvelle délinquance de masse ultraviolente et totalement désinhibée, qui n'a peur ni de la sanction ni de son exécution. Il va donc falloir faire face, si nous ne voulons pas que deux cents chasseurs vauclusiens aillent se faire justice comme ils en ont exprimé Monsieur le Premier ministre, pour faire face, nos concitoyens ne souhaitent ni discours ni bougies. Pour faire face, il n'est pas nécessaire de se lancer dans un énième concours Lépine de la nouvelle loi pénale, sans cesse réécrite sous le coup de l'émotion, et qui propose souvent des mesures déjà existantes, mais rarement appliquées. En effet, l'application des

du meurtre ignoble du commandant Éric Masson. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux l'ont également fait, hier, chez vous, en Avignon. J'adresse, bien sûr, à sa famille comme à ses collègues nos très sincères condoléances. Éric Masson est mort au cours d'une opération de lutte contre les trafics dans un point de en centre-ville d'Avignon. Dans le Vaucluse, tout particulièrement, la lutte contre le trafic de stupéfiants est l'une des priorités de l'action du Gouvernement. À ce titre, les opérations de sécurisation et de surveillance qui sont régulièrement menées dans les quartiers sensibles, notamment à Avignon et Carpentras, ont permis la découverte d'importantes quantités de produits stupéfiants, ainsi que d'armes à feu. L'engagement du ministère de l'intérieur dans cette lutte

Stéphanie Monfermé et Éric Masson sont tombés sous les coups de leurs agresseurs dans l'exercice de leur métier, créant un émoi dans la Nation tout entière. Le groupe Union Centriste veut s'associer à l'hommage qui leur a été rendu. Dans les rangs des forces de sécurité, au sein de la police nationale notamment, après les pleurs et la colère vient le temps des questions. Un grand malaise est perceptible. est vrai qu'il y a les mots dits, et ils ont été forts, monsieur le Premier ministre, dans les deux éloges funèbres que vous avez prononcés. Cependant, il y a aussi les mots qui sont écrits, ceux qui sont dans la loi, dans la loi pénale en particulier. Il y a surtout la force des décisions que nous attendons de la justice, qui doivent être fermes dans leur prononcé comme dans la réalité de leur application. Plus encore que ces mots, je crois que les policiers attendent de nous tous, mes chers collègues, nous qui représentons le peuple, une protection et un soutien encore plus forts. Monsieur le ministre, la loi pour une sécurité globale préservant nos libertés va entrer en vigueur et le Beauvau de la sécurité est en cours. Quelles décisions entendez-vous prendre pour rendre effectif, plus rapidement encore, le soutien que la Nation doit à ceux qui assurent notre sécurité quotidienne ?

en présence du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, le Premier ministre a rappelé son soutien plein et entier aux policiers. Il a également réaffirmé l'engagement du Gouvernement à concrétiser la volonté du Président de la République de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires au cours du quinquennat. Cet et mettra fin à la diminution des effectifs qui a été enregistrée depuis une dizaine d'années. Sur le plan budgétaire, les forces de sécurité intérieure (FSI) ont bénéficié d'une augmentation de 1,7 milliard d'euros de crédits depuis 2017, dont 137 millions d'euros supplémentaires pour l'immobilier, grâce au plan France Relance.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux du Beauvau de la sécurité qui ont été engagés par le ministre de l'intérieur, la question des réponses judiciaires et pénales fera l'objet d'une attention toute particulière, lors de la rencontre du 27 mai prochain. Enfin, le Premier ministre a également annoncé, mardi dernier, de nouvelles mesures fortes, qu'il s'agisse du plan de 10 millions d'euros pour sécuriser les commissariats et les casernes de gendarmerie, ou du renfort des moyens de la justice pénale grâce à l'engagement du garde des sceaux. En effet, il ne peut y avoir d'action policière efficace sans une réponse pénale dissuasive. Le Premier ministre a également annoncé vouloir inscrire dans la loi la limitation stricte des possibilités de réduction des peines. La peine de sûreté sera portée à trente ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme. Les violences contre les forces de sécurité intérieure seront désormais des délits délits spécifiques plus durement réprimés. Je pense notamment à la question des refus d'obtempérer. Enfin, le garde des sceaux prendra une circulaire demandant au parquet une fermeté stricte lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie, qui s'exercera par un défèrement systématique et un jugement rapide des auteurs. Je tiens à l'en remercier.

de la police nationale, témoigne dans la période singulière que nous vivons d'un nouveau cri d'alarme. Nous sommes nombreux au Sénat à l'avoir entendu, et nous serons certainement nombreux à soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de la protection des forces de l'ordre. Elles le méritent

républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le ministre des affaires étrangères, nous sommes des millions à être indignés par les images et les témoignages qui nous parviennent de Jérusalem : ratonnades, expropriations forcées de familles palestiniennes par des colons d'extrême droite, heurts ultraviolents et tirs meurtriers de l'armée israélienne sur l'esplanade et dans la mosquée Al-Aqsa, et maintenant bombardements de la bande de Gaza. Il y a déjà des dizaines de morts, des centaines de blessés. Ce qui est à l'oeuvre, c'est la colonisation systématique et illégale de Jérusalem-Est par le pouvoir extrémiste de Netanyahou, par une armée d'occupation, et par des colons fanatisés. L'ONU a rappelé que le déplacement forcé de civils par la puissance occupante était illégal au regard du droit international, et « pouvait s'apparenter à des crimes de guerre ». La procureure de la Cour pénale internationale parle de « fondement raisonnable » de crimes de guerre. Monsieur le ministre, que fait la France ? Notre voix, hier en première ligne, s'est éteinte au fil des ans. Vous avez enterré la résolution du Parlement pour la reconnaissance de l'État de Palestine. La démission internationale et la nôtre encouragent l'escalade meurtrière et colonisatrice de Netanyahou. Qu'attendez-vous pour réagir à ces violations graves et permanentes du droit international, à ces crimes de guerre établis et répétés, autrement que par des mots creux et par d'indignes renvois dos à dos du pouvoir criminel de Netanyahou et des victimes palestiniennes spoliées de leur droit à un État

que vous pratiquez comme une fuite en avant de nos responsabilités. Ce qui est en jeu, c'est Jérusalem-Est ! Vous savez très bien que c'est là le coeur de la crise. Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Sans sanction, Netanyahou ne bougera pas.

Ce texte est le fruit d'un travail de concertation que vous avez mené depuis plus de deux ans avec les élus locaux, et les aménagements proposés par le Gouvernement à travers la saisine rectificative vont assurément dans le bon sens. Permettez-moi de saluer la ténacité dont vous avez fait preuve dans ce dossier, madame la ministre, et la volonté forte de convergence que vous appelez de vos voeux, monsieur le président ! Nul ne conteste la nécessité ni la légitimité des objectifs qui ont inspiré cette loi.

Il ne vous aura pas échappé que les maires de France doivent encore faire face à un certain nombre de contradictions sur le terrain ... Ah ? Parmi elles, je citerai le raisonnement en pourcentage du nombre total de logements, qui a pour effet, tel le tonneau des Danaïdes, que plus vous construisez de logements, plus vous devez en produire. la difficulté de conjuguer un impératif de production importante avec celui de la « moindre consommation foncière » imposée par les documents d'urbanisme ; la contradiction manifeste entre le fait que les agglomérations disposent de plus en plus de compétences en matière de logement, mais que les exigences incombent toujours directement aux maires un taux de vacance des logements insuffisamment pris en compte sur les agglomérations dans leur globalité ; des constructions nouvelles qui se font au détriment de la rénovation de certains logements, alors que celle-ci est bien souvent mieux adaptée des infrastructures scolaires et périscolaires qui ne correspondent plus à la taille de la population ; un nombre d'agréments pas toujours en parfaite adéquation avec les demandes des communes, dont certaines voudraient faire plus Je pourrais poursuivre cette liste, mais je sais que les échanges que vous avez eus avec les élus locaux, durant ces derniers mois, vous ont permis d'entendre leurs craintes. Madame la ministre, pourriez-vous nous préciser les nouvelles dispositions du projet de loi 4D, introduites par la saisine rectificative ? Comment ? Comment entendez-vous poursuivre les relations constructives avec les élus sur cette question cruciale du logement aidé, ... Il faut conclure ! ... élus qui sont le plus à même de faire des propositions adaptées à leur territoire ?

Elle marquera, je crois, un tournant dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Je remercie le Sénat qui a tenu, hier, une conférence de presse. Monsieur le président, vous y étiez, accompagné des deux rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud,

la différenciation territoriale pour s'adapter aux réalités locales, de la décentralisation pour conforter les compétences des collectivités, de la déconcentration pour rapprocher l'État du terrain, et de la décomplexification, c'est-à-dire la simplification de l'action publique. Depuis sa version initiale, le texte a été enrichi, monsieur le sénateur, par une saisine rectificative qui vient notamment répondre aux préoccupations que vous soulignez sur le dispositif de la loi SRU. Les nouvelles mesures s'appuient largement sur le rapport du président de la commission nationale SRU, l'ancien sénateur Thierry Repentin. Elles ont été élaborées en concertation avec les acteurs du logement et les collectivités territoriales.

sachez que le régime d'exemption, notamment en matière de foncier ou de vacance, ainsi que l'intercommunalisation des objectifs font l'objet d'un travail continu, qui sera bien sûr poursuivi dans le débat parlementaire. Je suis certaine

et qui persistent : essoufflement, fatigue extrême, brouillard mental, difficultés de mémoire, douleurs articulaires, fourmillements, perte d'odorat, troubles du sommeil, tels sont certains des nombreux symptômes identifiés. Concrètement, les patients vivent une certaine forme d'errance médicale, alors qu'ils subissent un réel handicap, voire une perte d'autonomie. Savez-vous qu'il est parfois nécessaire de recourir à une rééducation respiratoire face à une respiration devenue dysfonctionnelle ? L'absence de reconnaissance, couplée aux conséquences sociales que représentent la perte d'emploi ou la vie de famille perturbée, ainsi que les incertitudes

est notre responsabilité du moment. Nous avons applaudi les soignants, salué leur engagement, loué leur dévouement. Et effectivement, nous leur en sommes tous tellement reconnaissants ! Désormais, il nous faut passer aux actes, car nombreux sont ceux, parmi eux, qui sont affectés par le covid long. Leur maladie n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Comment pouvons-nous les abandonner ainsi, alors qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts et qu'ils sont montés au front, sans hésitation, comme nous l'espérions ? Envisagez-vous, madame la ministre, de poser le principe d'une présomption de lien, dès lors que la maladie a été contractée par le soignant alors qu'il était en activité pendant la pandémie, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la reconnaissance légitime du covid long comme maladie professionnelle

au cours du temps. Aucun test biologique ne permet, à ce stade de l'affirmer ou de l'infirmer. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître ces formes de covid long. C'est chose faite depuis le 14 septembre 2020.

permanente au moins égal à 25 %. Ainsi, les formes graves, non respiratoires, de la covid peuvent être reconnues. En revanche, les formes bénignes des pathologies ne sont pas concernées et restent du ressort de la prise en charge des soins et des arrêts de travail, au titre de l'assurance maladie. En cas d'évolution, un nouvel examen est possible.

Ils font écho à une situation qu'on pensait suffisamment mise en lumière lors de cette crise du covid, mais qui hélas perdure ! Je parle, bien entendu, de la non-prise en compte de la revalorisation des salaires des soignants qui ne relèvent ni de la fonction publique hospitalière ni du secteur public.

hausse de la rémunération, c'est un statut qui est attendu. La demande de formation des personnels est également forte, dans un domaine où les crises de vocations dues aux conditions de travail ou à la concurrence des hôpitaux viennent peu à peu vider les établissements de leurs soignants. M. le ministre de la santé, le 27 janvier dernier, répondait en ces termes à ma collègue Guylène Pantel : « Nous garantirons une hausse des revenus à toute cette catégorie de personnes qui, de façon un peu aberrante effectivement, comme vous l'avez dit, n'ont pas bénéficié des revalorisations décidées dans le cadre du Ségur de la santé, mais qui travaillent aujourd'hui aux côtés des soignants madame la sénatrice, je peux vous l'assurer. » Tels étaient ses propos. ma question est simple : quelle réponse pouvez-vous leur apporter ?

de 160 euros par mois pour le secteur privé commercial. Elle est intégralement prise en charge, financièrement, par les pouvoirs publics. Le Premier ministre a demandé à Michel Laforcade, l'ancien directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, d'ouvrir des discussions pour étudier dans quelles conditions étendre le Ségur aux autres salariés du secteur médico-social que vous évoquez. Celles-ci sont en bonne voie. Par ailleurs, j'ai moi-même ouvert la porte pour que les aides à domicile intervenant chez les personnes âgées et handicapées de la branche d'aide à domicile bénéficient, à partir du 1 octobre 2021, d'une augmentation salariale de 13 % à 15 %.

Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. En mai 2019, son prédécesseur, Agnès Buzyn, promettait la prise en charge du deuxième accompagnant de tout enfant malade devant se déplacer sur le continent comme prestation légale. En novembre 2019, Josiane Chevalier, alors préfète de la Corse, confirmait cette intention, en annonçant la signature d'un décret au 1 janvier 2020. Consacrant cet engagement suprême, c'est en septembre de la même année que le Président de la République confirmait à son tour qu'une mesure entrerait en vigueur avant la fin du mois pour sanctuariser ce financement hors fonds d'action sociale. Voilà deux ans que votre Gouvernement a fait naître dans le coeur des enfants malades l'espoir de pouvoir bénéficier du droit à être accompagnés par leurs deux parents dans le difficile et courageux combat qu'ils mènent pour la vie. Deux ans de promesses faites aux associations, qui vaillamment portent la voix et la détresse de ces familles, pour mettre fin à une injustice connue et reconnue par votre Gouvernement. Deux ans au cours desquels vous allez de promesses en reculades, sans qu'une solution de financement pérenne soit aujourd'hui apportée. En attendant la parution de ce décret, promis maintes fois, mais toujours reporté, les frais de déplacement sont aujourd'hui pris en charge par un dispositif d'action sociale extra-légal temporaire des caisses primaires obligeant les parents à avancer les frais de déplacement. Pour ceux qui relèvent d'autres caisses, c'est la collectivité de Corse qui assure la prise en charge. Ce palliatif est fragile et nous ne pouvons nous en satisfaire à long terme.

la parole de l'État. Ma question sera donc simple, et la réponse que le Gouvernement apportera n'ira pas au parlementaire que je suis, mais s'adressera aux enfants malades et hospitalisés qui attendent que l'État honore sa parole et tienne ses promesses.

nous pouvons regretter que ce plan n'apporte aucun soutien à l'industrie européenne de défense. Il s'agit pourtant de l'un des secteurs essentiels à l'Union européenne. De nombreuses menaces pèsent sur notre continent. Sans industrie forte, l'autonomie stratégique est en péril, tout comme la sécurité de l'Union. Non seulement le plan de relance européen ne prévoit rien pour cette industrie, mais il a en plus été obtenu au prix d'une diminution du Fonds européen de défense, lequel passe de 13 milliards à 7 milliards d'euros pour les sept prochaines années, alors que de nombreux États dans le monde augmentent leur budget de défense. La crise de la covid-19 a ainsi souligné la nécessité de mettre en place

Par ailleurs, dans le cadre de son budget, la France doit travailler sans attendre à développer ses capacités stratégiques. Des mesures de soutien en faveur de l'industrie de la défense et de l'armement sont-elles prévues dans le plan de relance français ?

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le 4 mai dernier, une femme est morte sous les coups de son conjoint. Il a tiré dans ses jambes avant de l'immoler par le feu alors qu'elle était encore en vie. Cette femme s'appelait Chahinez Boutaa et elle avait trois enfants. Monsieur le Premier ministre, rien n'a été fait pour protéger cette femme, alors que tous les voyants étaient au rouge. Son mari avait été condamné à plusieurs reprises. Il possédait une arme. était sorti de prison en décembre 2020, sa femme avait de nouveau porté plainte en mars dernier. Malgré cela, Mme Boutaa n'avait pas de téléphone grave danger, son conjoint n'avait pas de bracelet anti-rapprochement et personne n'avait saisi son arme. En résumé, monsieur le Premier ministre, aucune des mesures que vous avez prises à la suite du Grenelle des violences conjugales conjugales n'a été mise en place pour cette femme. La mission d'inspection a rendu ses premières conclusions ce matin.

Monsieur le Premier ministre, tous les meurtres de femme ne peuvent pas être évités ; celui-là aurait dû l'être, si vous vous étiez donné les moyens d'appliquer des lois que vous avez vous-même votées. Ma question est donc simple : n'avez-vous pas honte d'une telle inefficacité de votre politique ?

Ce qui parfois me fait honte, c'est l'exploitation ... C'est l'exploitation cynique et obscène d'une situation que nous avons tous à déplorer avec beaucoup d'émotion

que nous n'aurons pas la main qui tremble si les dysfonctionnements sont avérés. Nous n'avons pas à avoir honte d'avoir fait ce que vous n'avez jamais fait

elles revendiquent régulièrement une meilleure prise en compte du reste à charge des AIS (allocations individuelles de solidarité), pour lesquelles l'Assemblée des départements de France (ADF) a engagé des négociations avec le Gouvernement, ces collectivités territoriales assurent et assument pleinement leurs missions. Comme le rappellent à juste titre nombre de leurs présidents et comme l'a démontré la crise sanitaire, les départements ne font pas de bruit, mais ils font le boulot C'est le cas pour la mise à l'abri et la protection des mineurs non accompagnés (MNA), puisque la compensation par l'État reste conditionnée à la signature d'une convention pour l'appui à l'évaluation de la minorité

de ces jeunes, qui ont brillamment réussi leur parcours d'insertion et d'intégration, ne se fasse souvent qu'à la faveur d'une forte mobilisation de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle une proposition de loi tendant à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) a été déposée par Jérôme Durain et plusieurs de nos collègues. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer votre position quant à la prise en charge effective par l'État de l'accueil d'urgence de ces jeunes, ainsi que sur les mesures qui pourraient être retenues, à destination des préfectures, afin d'assouplir la régularisation lorsque l'employeur atteste de la qualité professionnelle et de la parfaite

le 17 mai 2018 entre le Gouvernement et l'Assemblée des départements de France, avec un volet financier opérationnel. Un financement exceptionnel à destination des départements

pour contribuer à l'identification des étrangers qui se déclarent MNA. Enfin, plusieurs actions ont été engagées pour limiter les ruptures de droits au passage de la majorité. Nous sécurisons donc la phase d'évaluation de la minorité pour que les vrais mineurs puissent faire l'objet d'un placement à l'ASE et nous proposons à ceux d'entre eux qui, placés à l'ASE, sont engagés dans un parcours

actes d'état civil. À l'occasion de son déplacement dans le Pas-de-Calais en janvier 2018, le Président de la République a voulu renforcer ce dispositif par la mise en place additionnelle d'une prestation d'aide alimentaire, qui représente 1 800 repas distribués

Napoléon I, dont le Président de la République commémorait, le 5 mai dernier, le bicentenaire de la mort. Deux cents ans plus tard, nous saluons toujours la création des préfectures, premier pas vers la déconcentration. ministre, dès le lendemain de cette commémoration, vous annonciez devant l'ensemble des préfets et sous-préfets la fin de ce corps d'État. Cette fonctionnalisation des préfets est incompréhensible. Elle est incompréhensible, car elle déconstruit l'État et son autorité, une autorité plus que jamais essentielle en ces temps troublés par l'insécurité, la violence et les différentes crises que nous subissons. Elle est incompréhensible, car elle rompt le lien de proximité entre l'État et les territoires, une proximité qui est la clé de voûte de l'action de l'État déconcentré- le couple préfet-maire a démontré toute son efficacité depuis le début de la crise sanitaire. Représentants de l'État dans les territoires, les préfets ne sont pas de simples administrateurs. Ils sont le lien entre l'État et les élus locaux.

Car, sans déconcentration, il n'y aura ni différenciation, ni décomplexification, et encore moins de décentralisation ! Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous affirmer, ici, au Sénat, que le corps préfectoral ne disparaîtra pas ? Pouvez-vous nous assurer que cette réforme n'ouvre pas la porte à l'arbitraire dans la fonction publique ?

Vous avez devant vous un Premier ministre qui a eu l'immense honneur d'être secrétaire général de préfecture et sous-préfet d'arrondissement chef-lieu dans sa vie professionnelle- un vrai bonheur !

? Dois-je vous rappeler que mon Gouvernement a placé les préfets aux avant-postes d'un des axes essentiels de la politique de l'État pour le pays, à savoir

loin de porter atteinte à ces éminentes et indispensables fonctions, vise au contraire, non seulement à les conforter,

Ce n'est pas là la marque d'une gestion des ressources humaines moderne et dynamique. Nous allons donc revaloriser ce beau métier, cet indispensable métier,

en matière de ressources humaines et de gestion budgétaire, tout en déconcentrant des crédits depuis Paris. Dans la loi de finances pour 2021, texte examiné dans cette assemblée, l'essentiel des effectifs nets de l'État, hors éducation nationale, a été créé dans les échelons déconcentrés. Nous allons évidemment instaurer une filière de la préfectorale, car celle-ci suppose expérience, parangonnage, compétences spécifiques. Ce n'est pas parce que, fidèles à l'ordonnance de 1945, nous allons redonner toute sa place à l'interministérialité de la haute fonction publique

trop dilué ... Nous devons le rassembler autour de l'autorité préfectorale. Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'à l'heure actuelle, hors éducation nationale, 85

nationale d'administration (ENA), seront donc affectés dans leur premier poste sur des fonctions opérationnelles. Aucun ne rejoindra plus les fonctions de contrôle des grands corps de l'État ou des fonctions juridictionnelles. Priorité au terrain ! L'administration préfectorale, je vous le dis, sera restaurée dans son prestige- il est déjà immense -et renforcée dans ses attributions et dans le beau métier qu'elle représente.

Madame la ministre, ayant été maire durant des décennies, vous savez à quel point les travaux de rénovation de voirie sont une constante dans la vie municipale. Or, aujourd'hui, nombre de communes n'ont plus les moyens de financer ces travaux, deux raisons essentielles. D'une part, le département et la région, qui traditionnellement aidaient le plus les communes à effectuer ces travaux, se sont appauvris. D'autre part, l'État a puissamment réorienté ses priorités avec le plan de relance et la transition écologique. on a mis la voirie municipale et sa sécurisation de côté, comme s'il s'agissait d'une sous-dépense, une dépense d'un autre temps, en marge du progrès. C'est absurde il ne peut y avoir de relance ni de transition énergétique sans voirie municipale. Pas de voiture électrique ou à hydrogène sans routes à emprunter ! Pas de plan Vélo sans requalification des voies ! Et il est question ici non pas du simple entretien,

C'est une excellente décision, que nous attendions tous, avec, de surcroît, un engagement sur cinq ans. Permettez-moi tout de même de signaler que cette progression est très disparate selon les territoires : 30 % à Paris, 14 % à Lyon, 7 % à Saint-Étienne. Il faudra nous expliquer cette inégalité de traitement. Je tiens surtout à vous interpeller sur la situation des étudiants inscrits en parcours accès santé spécifique (PASS), très pénalisés en cette année de transition par la réforme des études de santé.

Quelle injustice pour les étudiants de première année de PASS ! Imaginez leur déception d'être dans cette année de transition si défavorable, sans augmentation du nombre d'admis, après avoir subi une année si difficile en raison du confinement.

En dépit de leur mobilisation auprès des pouvoirs publics ces derniers mois, rien ne semble avoir été fait pour anticiper cette situation. Elles connaissent en effet les plus grandes difficultés à s'approvisionner en bois et dérivés de bois, polyuréthane, polystyrène et plaques de plâtre, pour ne citer que quelques exemples. Les prix de l'acier et du PVC ont augmenté respectivement de 106 % et de 114 %, celui du cuivre de 51 %. Tout le paradoxe est là : les demandes des particuliers et la commande publique en matière de construction sont en hausse, mais les entreprises risquent de ne pas pouvoir les satisfaire faute d'approvisionnements corrects. Ces pénuries entraînent déjà l'arrêt de certains chantiers. Elles vont certainement affecter de nombreux corps de métiers en conséquence, dans un contexte de relance économique et de préservation impérative de l'emploi.

Le cas du bois est révélateur : depuis plusieurs années, les grumes françaises, le chêne en particulier, sont massivement exportées vers l'Asie et la Chine, à un prix supérieur de 25 % à 30 % à ce que les scieries françaises sont en mesure de proposer, pour être ensuite importées- si la Chine le veut bien ! -une fois transformées. Les professionnels de la filière bois ont pourtant maintes fois alerté sur le manque croissant de matières premières pour les transformateurs locaux, sans être pour autant entendus. Aujourd'hui, nous en voyons le résultat : c'est tout le tissu manufacturier français qui est menacé et, une fois de plus, cette situation met fortement en cause notre souveraineté industrielle. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour garantir cette autonomie nécessaire au bon fonctionnement

Nous pourrions y ajouter l'augmentation du prix du baril de pétrole, qui se traduit à la fois par une hausse des prix de revient pour les secteurs énergivores et par une augmentation du prix de production des matières plastiques, avec des difficultés identiques à celles que vous avez évoquées.

les transports et les échanges en activant un certain nombre de mesures douanières ; en menant des actions diplomatiques auprès des pays concernés ; ou encore en réunissant les filières, pour les inciter à mutualiser un certain nombre de moyens et à dissuader les plus grands donneurs d'ordre de constituer des stocks de précaution qui priveraient de plus petits acheteurs.

nous en sommes tous conscients : nous ne pourrons organiser les festivals pendant l'été qu'à la condition de les préparer en amont, avec la kyrielle de mesures qui devront s'imposer à juste titre. Petit à petit, vous desserrez l'étau : vous levez certaines contraintes, mais globalement les festivaliers sont face à trop d'inconnues, alors que les dates se rapprochent.

Au mois de septembre, dans les Ardennes, se tient le festival mondial des théâtres de marionnettes : ses organisateurs sont très inquiets, car certains festivals sont reprogrammés plus tard dans l'été, ce qui va provoquer une concentration des événements culturels. La mutualisation habituelle du matériel va être mise à mal du fait du resserrement des dates des festivals. La question du passe sanitaire illustre tout à fait le questionnement que je formule devant vous aujourd'hui. Comment organiser efficacement les contrôles ? Comment appliquer la jauge des quatre mètres carrés par personne ? Comment s'adapter au mieux à toutes les situations ? Comment encadrer la circulation des foules ? Comment sera réglée la question des buvettes ? Les festivaliers ont besoin de connaître l'état de la réflexion au sein du ministère. Sur d'autres problématiques liées à la covid, l'état d'impréparation du Gouvernement n'a pas aidé à atteindre les objectifs fixés. Je compte sur vous pour nous éclairer au sujet de la culture. Madame la ministre, je pense, j'espère que vous allez être meilleure que les autres. Ma question est simple : quelles garanties le Gouvernement compte-t-il donner pour les festivals de l'été ?

prochain en Amérique, le 30 mai dans le reste du monde, se tiendront les élections consulaires pour élire les conseillers des Français de l'étranger et les délégués consulaires. Les électeurs auront également la possibilité de voter par internet du 21 au 25 mai. C'est heureux et, compte tenu des conditions sanitaires, j'encourage tous nos compatriotes à l'étranger à choisir ce mode de vote pour s'exprimer. Il y a deux jours, nous avons appris par le le dépôt à l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement au projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. permettre, dans les circonscriptions où le scrutin poserait difficulté, le report des élections consulaires. Compte tenu des circonstances auxquelles certains pays font face, on peut comprendre que le vote à l'urne puisse être difficile, voire impossible.

À neuf jours de l'ouverture du scrutin par internet et à dix-sept ou dix-huit jours du vote à l'urne, je souhaite lutter contre les fausses nouvelles et mobiliser les électeurs à l'étranger pour les inciter à participer aux élections consulaires. Pouvez-vous nous indiquer la liste des circonscriptions concernées par un report éventuel afin de clarifier la situation, alors que nous nous engageons dans la dernière ligne droite ? À défaut, nous souhaitons savoir combien de circonscriptions sont susceptibles d'être affectées et à quelle date leur liste sera connue ! La parole

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Conformément à l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Elles seront ratifiées

qui vient de se terminer, parce que je participais à une réunion entre le Président de la République, Emmanuel Macron, et le Président de la République argentine. Au cours de cette séance, M. Pierre Laurent a interrogé le Gouvernement sur la situation au Proche-Orient et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne lui a répondu. Je voudrais dire fortement combien je suis très préoccupé par la gravité de la situation au Proche-Orient. Cette situation, chacun le sait, résulte d'une absence de perspectives politiques. Elle n'a que trop duré et ne pourra que continuer à produire des souffrances et de la violence si la volonté n'est pas là d'avancer résolument vers l'établissement de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, avec Jérusalem pour capitale. Depuis plusieurs jours, particulièrement cette nuit, et encore en ce moment, les affrontements s'intensifient, et le bilan est déjà très lourd parmi les civils palestiniens et israéliens. Le cycle des violences en cours à Gaza, à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie et dans plusieurs villes d'Israël risque de conduire à une escalade majeure. En moins de quinze ans, la bande de Gaza a connu trois conflits meurtriers. Tout doit être fait pour en éviter un quatrième. Il est donc absolument indispensable que tous les acteurs, sans exception, fassent preuve de la plus grande retenue et s'abstiennent de toute provocation et de toute incitation à la haine pour mettre un terme à des violences dont les premières victimes sont les populations civiles palestiniennes et israéliennes. Pour ces populations, comme pour toute la région, la seule priorité, à cette heure, doit être l'apaisement des tensions. Je m'entretiendrai très prochainement avec mes homologues israélien et palestinien pour leur faire passer l'ensemble de ces messages et pour contribuer à la désescalade. Je vais aussi m'entretenir dans quelques heures avec mon homologue égyptien pour coordonner nos démarches avec les efforts de l'Égypte, que je salue, qui travaille en ce moment même à un retour au cessez-le-feu à Gaza. retour au cessez-le-feu à Gaza. La France condamne dans les termes les plus fermes les tirs de roquettes et de missiles qui se sont intensifiés depuis la bande de Gaza et ont visé Jérusalem et plusieurs zones habitées du territoire israélien, y compris Tel-Aviv. Ces tirs risquent désormais de provoquer un nouveau cycle d'affrontements. Effectués en violation du droit international et revendiqués par le Hamas, ils ne sont pas acceptables. Nous sommes aussi gravement préoccupés par la situation à Jérusalem. La stricte préservation du historique sur l'esplanade des mosquées est indispensable ; j'ai abordé cette question avec mon homologue jordanien, compte tenu du rôle spécifique reconnu à la Jordanie sur les lieux saints de Jérusalem. Je rappelle également notre totale condamnation de la colonisation, qui est contraire au droit international. Les menaces d'évictions forcées visant des résidents palestiniens de Jérusalem-Est à proximité de la vieille ville, notamment à Cheikh Jarrah, participent à l'entreprise de colonisation et alimentent les tensions. Enfin, le droit à manifester pacifiquement doit être garanti.

tensions. Nous n'avons qu'un seul objectif : une reprise du dialogue entre les parties, en vue d'une résolution juste et durable du conflit dans le cadre du droit international,

est à Mme Claudine Lepage. Cet amendement vise à rappeler les cadres que la France s'est engagée à respecter en mentionnant les ODD et la stratégie Droits humains et développement de 2019. La stratégie Droits humains et développement a pour ambition de formaliser le cadre de l'action française d'appui au respect, à la protection et à la réalisation des droits humains la coopération. Conformément au nouveau consensus européen pour le développement, elle vise également à intégrer l'approche fondée sur les droits humains dans l'ensemble des actions de coopération au développement menées par la France. Le développement crée les conditions de jouissance effective des droits humains pour toutes et tous, et le respect de ces droits participe à un développement véritablement durable. Ainsi, il s'agit de continuer à faire évoluer l'approche française, en ne concevant plus les programmes de développement seulement comme des actions de solidarité, mais également comme des outils de soutien à la mise en oeuvre des obligations internationales des États en matière de droits humains. Si la réalisation des droits humains est l'idéal commun à atteindre, c'est également le moyen de parvenir à un développement durable.

En effet, le fonds dédié du groupe de travail pour l'agenda sur l'identité juridique des Nations unies, auquel il est ici fait référence, n'a pas encore été créé, car le montant minimum requis de 5 millions de dollars américains n'a pas été atteint. En attendant, le groupe RDPI appelle la France à continuer à soutenir les agences onusiennes qui travaillent dans ce groupe. L'enregistrement des naissances et l'identité juridique des enfants sont

sans identité, ces enfants n'ont pas accès à la justice. Notre inquiétude est d'autant plus grande que les taux d'enregistrement des enfants en Afrique risquent de reculer pendant la pandémie de covid-19. C'est pourquoi nous soutenons vivement la campagne lancée en juin 2020 par l'Union africaine et l'Unicef, intitulée « Mon nom est personne », ce qui rappelle un titre de de film célèbre. Cette initiative vise à rallier les États membres de l'Union africaine autour d'un engagement en faveur de l'enregistrement universel des naissances pour tous les enfants en 2030. Je tiens à saluer le travail remarquable des fonctionnaires d'état civil de nos collectivités qui, dans le cadre de la coopération décentralisée, participent

le PNUD et le département des affaires économiques et sociales de l'ONU s'est constitué ; des États comme la Grande-Bretagne, la Suisse ou le Canada ont déjà répondu présents à cette participation, sur la

La participation de tous à l'élaboration des politiques publiques les concernant est un enjeu majeur de demain. Les femmes sont particulièrement mises à l'écart dans les instances de décision ; cet amendement vise donc à ce que notre aide publique au développement les considère comme des décisionnaires et les encourage à concourir aux politiques publiques qui les concernent. Je ne développerai pas plus avant cet argumentaire, qui est le même que pour l'amendement n° 207, lequel avait été satisfait par l'adoption de l'amendement n° 1 rectifié de Mme Doineau.

par les droits humains en général et non à l'égalité entre les femmes et les hommes ni à la participation des populations à la politique de développement durable, traitées à d'autres endroits du texte. Cela ne nous semble pas approprié : l'avis est défavorable.

Vulnérables parmi les vulnérables, les filles sont doublement discriminées du fait de leur sexe et de leur âge et se trouvent encore trop souvent négligées sur le plan de la santé, de l'éducation, de la nutrition et de la protection. Une mobilisation forte et marquée est donc indispensable. Il est important que la conception de l'égalité diffusée par notre aide publique au développement s'applique dès la naissance. naissance. La loi de 2014 actait ainsi l'importance de la prise en compte de la situation spécifique des filles par l'intégration de leurs besoins et de leurs droits dans la définition et la mise en oeuvre des actions de solidarité internationale. Cet aspect revêt une importance majeure dans les pays définis comme prioritaires pour la France, où les moins de 18 ans constituent généralement la moitié de la population.

À l'instar de la loi de 2014, cet amendement vise à assurer une visibilisation de ce problème particulier.

monsieur le ministre,

Mme Claudine Lepage. Dans ce projet de loi, les mutilations sexuelles sont considérées comme étant liées à la santé ou encore à l'égalité entre les filles et les garçons. Or il est nécessaire d'affirmer qu'elles relèvent des droits humains. Cet amendement tend donc à insérer une mention des mutilations sexuelles dans le paragraphe relatif aux droits humains.

? L'alinéa 63 présente l'approche de la France en matière de droits humains : État de droit, identité juridique, liberté d'expression et de croyance, dépénalisation de l'homosexualité, protection de l'enfance, etc.

contre la haine et les discriminations anti-LGBT+. Dans le cadre de ce plan, des engagements ont été pris en matière de politique internationale, parmi lesquels une amplification de l'action de la France en faveur de la défense des libertés fondamentales des personnes LGBT+, partout dans le monde.

? Les principes de Yogyakarta sont « des principes sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre ». Ils ont été présentés le 26 mars 2007 au Conseil des droits de l'homme, puis le 7 novembre de la même année lors d'un événement en marge de l'Assemblée générale des Nations unies coorganisé par l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Ces principes, élaborés au nom d'une coalition d'ONG, n'ont pas de valeur contraignante en droit international des droits de l'homme et ils n'ont pas été

Je me suis déjà exprimé sur ce sujet pour rappeler que les principes de Yogyakarta, dont je partage complètement

M. Lucien Stanzione. Cet amendement vise à intégrer la question de l'extrême pauvreté dans l'approche fondée sur les droits humains et à renforcer les capacités des citoyens afin qu'ils soient en mesure de faire valoir leurs droits. des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, adoptés en septembre 2012 par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies avec le soutien de la diplomatie française, constituent une avancée majeure dans la pensée sur l'extrême pauvreté en tant que grave violation de l'ensemble des droits de l'homme et sur les politiques pour l'éradiquer, consacrant ainsi l'approche par les droits. Ces principes Ces principes constituent un instrument permettant aux pays comme aux organisations internationales de veiller à ce que les politiques publiques, y compris les efforts d'éradication de la pauvreté, atteignent les membres les plus pauvres de la société, respectant et défendant leurs droits, et tiennent compte des importants obstacles sociaux, culturels, économiques et structurels à l'exercice des droits de l'homme auxquels les personnes vivant dans la pauvreté se heurtent. Par ailleurs, ainsi que le souligne ATD Quart Monde, ces principes directeurs identifient explicitement les démarches que les gouvernements et les acteurs concernés devraient entreprendre pour garantir que toute personne puisse jouir de ces droits et que la misère soit éradiquée. Cet amendement tend donc à introduire une continuité des engagements pris par la France sur la scène internationale.

et les droits de l'homme soient également intégrés dans le projet de loi et servent d'éléments structurants ». L'introduction de cette référence à l'alinéa 63 nous semble donc essentielle.

C'est regrettable pour cette organisation, qui joue un rôle central dans la lutte contre l'extrême pauvreté.

Il apparaît toutefois que la mention de la convention internationale des droits de l'enfant dans le paragraphe sur l'approche par les droits gagnerait à être suivie de la mention des quatre principes directeurs que sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit à la participation, afin de renforcer la visibilité de la convention internationale des droits de l'enfant dans ce projet de loi, qui en fait désormais une priorité.

tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouvent des millions d'enfants dans le monde, renforcer la visibilité de la convention internationale des droits de l'enfant dans ce projet de loi et en préciser les priorités permettrait d'effectuer un cadrage plus clair des missions des politiques publiques françaises. Il ne s'agit pas d'un ajout superflu, mais bien de la marque de l'engagement de la France en faveur de la protection des droits de l'enfant et d'une garantie de la prise en compte de leurs droits et de leur situation particulière de vulnérabilité. La

et les ressources, et parfois même leur culture, ont augmenté de façon spectaculaire. Aujourd'hui, ces défenseurs ne jouissent pratiquement d'aucune reconnaissance juridique

Pour autant, nous soutenons clairement ces populations. Leurs défenseurs sont des hommes et des femmes qui luttent pour que ces populations ne soient pas dépossédées de leurs terres ou déplacées. Ils luttent aussi

s'agissant des territoires où vivent des peuples autochtones. Monsieur le ministre, je rappelle que la France est signataire de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007. Par ailleurs, lors de la visite du chef Raoni, le 16 mai 2019, l'Élysée a indiqué que la France défend les droits des autochtones, notamment en tant qu'acteurs essentiels de la préservation des forêts et de la biodiversité et, par conséquent, engagés dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Les auteurs de cet amendement soulignent précisément ce lien entre peuples autochtones et protection de l'environnement. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

Carlotti. Nous souhaitons que la France prenne en compte l'exigence de responsabilité sociétale des acteurs, publics ou privés, et qu'elle la promeuve auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Pour cela, il sera demandé à nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, d'exercer un devoir de vigilance quant à leur attitude à l'étranger, de respecter les droits humains, environnementaux et sociaux et, bien sûr, de maîtriser leur impact. Tel est le sens de cet amendement. Au demeurant,

Le Gouvernement a accepté un autre amendement tendant à introduire une référence au principe « ne laisser personne de côté » consacré dans l'agenda 2030 fixant les ODD.

comme bien public mondial. La promotion de la santé comme bien public mondial « est » bel et bien un élément constitutif et même une priorité de la politique française de développement. J'en citerai quelques exemples : les 10 millions d'euros annuels donnés au Fonds français Muskoka, dont l'objectif est d'améliorer l'accès des femmes à des soins de santé de qualité en Afrique, nos contributions aux fonds multilatéraux, notre contribution de 2 millions d'euros à l'Académie de la santé de l'OMS, située à Lyon, ou l'initiative Santé en commun de l'AFD.

: La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret. La pandémie que nous traversons a démontré l'importance de bénéficier d'un système de santé solide. Elle nous a fait redouter le scénario du pire pour les pays en développement, notamment les pays de l'Afrique subsaharienne, dont les systèmes de santé sont très fragiles et manquent cruellement d'investissements. cette pandémie n'est pas terminée. De nouvelles crises sanitaires mondiales ne sont malheureusement pas exclues à l'avenir. Dans ces pays en développement, plus particulièrement africains, les défis sanitaires sont le lot du quotidien. Après soixante ans de politiques d'aide au développement dans de nombreux pays classés comme prioritaires, les infrastructures sanitaires demeurent défaillantes et parfois même absentes. Les personnels de santé sont en nombre insuffisant, l'absence de médicaments engendre le commerce illégal sur les marchés et l'absence d'assurance maladie empêche les plus précaires de se soigner.

brute française a été allouée au secteur de la santé, ce qui est très peu. Il est temps de s'attacher aux effets sur le terrain. C'est pourquoi cet amendement vise à contribuer au renforcement des systèmes de santé de base des pays en développement qui ne sont pas soutenus par les programmes internationaux, concentrés sur les programmes mondiaux de lutte contre les épidémies et les urgences sanitaires. Il tend d'abord à agir prioritairement au bénéfice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes dans le cadre des droits à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les enfants. enfants. Il vise ensuite à assurer la disponibilité de médicaments en qualité et quantité suffisantes sur tout le territoire pour les pathologies à traiter. Enfin, il a pour objet de consolider globalement les systèmes de santé en renforçant la formation des personnels de santé et en accompagnant les États dans la réforme de l'organisation et du financement de leurs systèmes.

la crise sanitaire a jeté une lumière crue sur les inégalités en matière sanitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique abrite un quart des personnes malades dans le monde, mais ne fabrique qu'une part infime- moins de 2 % -des médicaments consommés sur le continent. Cet amendement vise donc à permettre aux pays en développement d'acquérir leur autonomie dans le domaine de la recherche, en particulier sanitaire. Cet objectif ne pourra être atteint qu'en renforçant la coopération entre les chercheurs et en favorisant la création de laboratoires implantés localement. Cela permettrait à ces pays de mener des travaux de recherche innovants et de pouvoir faire face aux crises épidémiques qui les touchent plus localement. Mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement afin de faire vivre la solidarité et de doter les pays en développement de leviers à même de leur octroyer un véritable pouvoir d'action dans le domaine de la recherche. L'adoption de cet amendement aura aussi pour effet d'enrayer la fuite des cerveaux et de permettre aux chercheurs de ne pas avoir à s'expatrier pour des raisons professionnelles.

La seule levée des brevets n'est pas suffisante pour compenser les inégalités vertigineuses d'accès aux vaccins. Elle est toutefois nécessaire pour démultiplier les capacités de production de doses. On peut saluer le fait que la France envoie en Afrique de l'Ouest un demi-million de doses de vaccins

qui consacre les vaccins comme biens publics mondiaux et permette la levée des brevets.

il est mort

afin d'aider les pays à atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé d'ici à 2030.

Dans son discours de Ouagadougou de novembre 2017, le Président de la République a affirmé que le sport constitue un « levier d'action

l'insertion socio-économique, laquelle désigne un processus conduisant à l'insertion d'une personne dans son milieu social et dans un milieu de travail. Trouver un emploi requiert une adaptation au milieu dans lequel on vit et une maîtrise des méthodes de recherche et d'obtention d'un emploi. emploi. De nombreux facteurs interdépendants influent sur l'insertion réussie, qui se traduit par une intégration satisfaisante, tant pour la personne que pour la société. Ces facteurs, tant sociologiques qu'économiques, politiques, culturels, démographiques et géographiques, ne doivent pas être négligés. cet amendement proposent donc de prendre en compte l'employabilité à travers le défi global que représente l'insertion socio-économique des populations.

au niveau mondial. La covid-19 va donc encore aggraver le déficit de financement annuel de l'éducation dans les pays les plus pauvres, évalué à 200 milliards de dollars par an. Si des engagements ne sont pas pris, avec une programmation financière précise et adéquate, les risques de voir une génération entière sacrifiée demeurent immenses, notamment dans les pays les plus pauvres. Pour ces raisons, nous proposons de mettre l'accent sur l'éducation. Quel est l'avis de la commission

Est-ce la misère qui les pousse à s'enrôler ? » Le Président Bazoum lui a répondu : « Je tiens à affirmer qu'il n'y a pas un lien direct, de cause à effet, entre la pauvreté et le terrorisme. C'est surtout le manque d'éducation, par l'école, qui explique l'enrôlement de certains jeunes. » Tout est dit

En effet, l'éducation est le gage d'un développement durable en mesure d'apporter des effets concrets face aux défis socio-économiques, politiques et démographiques auxquels les pays en voie de développement sont confrontés. sont confrontés. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'accès à l'éducation est un objectif prioritaire ; mais, dans les faits, et bien que la France consacre 992 millions d'euros d'aide bilatérale à l'éducation dans les pays en développement, seulement 1,8 % de l'APD bilatérale est allouée à l'éducation de base et 19 % de ces fonds sont attribués aux pays les plus fragiles classés comme étant prioritaires. À titre d'exemple, seulement 5 % de l'APD bilatérale allouée à l'éducation de base est orientée vers les pays du Sahel, alors même que ces pays se trouvent à la croisée de tous les défis du développement. Le surpeuplement des classes, le nombre réduit d'enseignants travaillant dans des conditions peu valorisantes et faiblement rémunérés par les États, l'insuffisance de manuels scolaires adaptés et actualisés, le délabrement des infrastructures ou l'obsolescence des équipements ont pour conséquence de dégrader les conditions d'études. les conditions d'études. Le présent amendement vise donc à aboutir à une meilleure répartition des crédits de l'aide publique au développement en faveur de l'éducation en les orientant vers le financement des infrastructures et des équipements scolaires. Ces disparités sont également liées au lieu de résidence, puisque les zones rurales défavorisées bénéficient peu, sinon quasiment pas, d'initiatives publiques en faveur du développement. C'est pourquoi cet amendement tend à insister sur la nécessité de couvrir de manière uniforme l'ensemble des territoires ruraux et urbains., urbains., ces insuffisances entravent l'effort d'un système éducatif inclusif et performant. Pourtant, il y a urgence. En effet, selon l'Unicef, en 2030, le nombre d'enfants à scolariser atteindra 619 millions, dont 444 millions pour la seule Afrique subsaharienne. Ces enfants sont la force vive qui prendra part demain au développement de leur pays. Mes chers collègues, en adoptant cet amendement pour renforcer la qualité des conditions d'études, nous ferions le choix, je le crois, d'une politique d'aide au développement responsable, qui agit à la racine des causes premières des inégalités telles que l'analphabétisme, la déscolarisation et la fuite des forces vives vers les pays du Nord.

qui a lancé la refondation du programme d'enseignement des mathématiques au collège. Des enseignants maliens, avec l'aide des enseignants de mathématiques français du lycée français, se sont engagés dans

Pourtant, nombre de ces jeunes sont privés d'emploi et ne bénéficient d'aucune perspective, ce qui constitue un véritable frein pour l'effort d'un développement économique et social. L'autre conséquence est que ces jeunes nourrissent les flux migratoires vers les pays du Nord, deviennent des proies privilégiées pour les passeurs et sont parfois même recrutés par des groupuscules groupuscules terroristes. À cet égard, le cas des pays du Sahel est éloquent. C'est donc à ce niveau que notre aide publique au développement doit obtenir des résultats concrets, favorisant l'employabilité de ces jeunes. Or les économies des pays en développement, plus particulièrement celles de la bande sahélo-saharienne, sont marquées par une inadéquation entre la formation et l'employabilité. En effet, les formations dispensées dans des domaines divers tels que le commerce, le droit, l'économie, les finances et les ressources humaines occupent une place prépondérante et produisent un nombre important de citadins intellectuels, finalement touchés par un chômage massif., massif., les secteurs primaire et secondaire offrent davantage de débouchés, permettent une insertion plus rapide à l'aune des besoins de ces populations et constituent une voie privilégiée pour relever les défis de l'essor de l'industrialisation et, par exemple, de la modernisation de l'agriculture sous-régionale. La valorisation de ces secteurs nécessiterait la mise en place et le renforcement de filières d'enseignement technique industriel et d'enseignement agricole. Par ailleurs, l'existence d'une main-d'oeuvre qualifiée est une condition permettant l'accueil de capitaux en vue des investissements nécessaires dans la transformation locale des produits. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.

totale à l'éducation et 50 % de cette APD éducation à l'enseignement de base dans les pays à faible revenu et les États fragiles, avec une priorité pour les pays d'Afrique subsaharienne.

Dans son discours de Ouagadougou, le Président de la République a déclaré : « Renforcer vos établissements et vos cursus universitaires, c'est multiplier les partenariats, les échanges, les formations croisées, les doubles diplômes, qui répondront à vos attentes. » Campus France attentes. » Campus France porte notamment le programme « Partenariats avec l'enseignement africain », aux côtés du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Cet appel à projets financé par l'AFD, qui est l'un des volets de la stratégie « Bienvenue en France », vise à financer

d'une anecdote. Il y a une dizaine d'années, dans le cadre d'une mission parlementaire, je me suis rendu dans l'un des pays les plus pauvres d'Amérique centrale, le Salvador, pays qui doit faire face à de nombreuses difficultés, notamment liées à une insécurité chronique.

coorganisé, pour la première fois, une table ronde intitulée « Investir dans le sport pour les ODD ». Cet événement avait pour objectif de réfléchir à des politiques et des initiatives concrètes visant à renforcer la contribution du sport et des investissements qui y sont liés à l'atteinte des objectifs de développement durable. Quant à l'Agence française de développement, elle déploie une stratégie appelée « Sport et développement », qui fait du sport l'un des nouveaux axes de son action, en mettant l'accent sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Partout et de tout temps, le sport est un vecteur d'émancipation et d'expression. Sa pratique permet d'inculquer des valeurs essentielles, notamment aux jeunes. Il est alors primordial d'inscrire dans la loi que la France fera la promotion du sport, qui est un outil réel d'inclusion sociale, d'égalité entre filles et garçons et, naturellement, un instrument de promotion de la paix. Quel

a permis l'adoption d'un langage plus robuste sur les droits de l'enfant- je m'en félicite -, y compris sur l'indispensable approche multisectorielle de l'enfance, notamment grâce aux mentions des droits de l'enfant et de la convention Pour cette raison, il semble souhaitable et logique de préciser que la France soutient l'Unicef, certes sur l'éducation, qui est déjà une priorité affirmée dans la loi, mais également dans son approche multisectorielle pour l'effectivité des droits de l'enfant.

afin d'encourager les États partenaires à favoriser les systèmes scolaires publics, inclusifs, stables, bien financés, gratuits et conformes aux droits humains. faire en sorte que l'école dans ces pays soit, comme l'école publique chez nous, un sanctuaire préservé des intérêts marchands et, bien sûr- nous l'avons tous en tête -des financements religieux et des influences qui vont avec.

Merci,

une révision du tableau des prévisions d'APD figurant dans le rapport annexé, qui présente pour la première fois la trajectoire globale de notre APD, conformément à l'engagement pris par le Président de la République. Ce tableau repose

Une nouvelle fois, l'enjeu est non pas de dire que la France ne doit plus accueillir de jeunes étrangers en formation, mais de savoir dans quelle mesure il s'agit d'aide publique au développement. Cette comptabilisation pose en effet deux questions. Premièrement, si la France apporte effectivement presque 1 milliard d'euros au secteur de l'éducation dans le cadre de son APD, la grande majorité de cette somme, soit environ 70 %, est versée au titre des frais d'écolage. signifie que 70 % de cette somme ne quitte jamais le territoire français et n'est pas dirigée vers le renforcement des systèmes éducatifs locaux. Deuxièmement, cela crée des situations paradoxales. Ainsi, les frais d'écolage des étudiants chinois représentent chaque année 67 millions d'euros, comptabilisés dans l'aide publique au développement française. Au total, un peu plus de 15 % des frais d'écolage sont alloués aux pays prioritaires de l'aide française. Ce déséquilibre risque encore d'augmenter dans les années à venir à la suite de la mise en place du plan « Bienvenue en France », qui nécessitera une augmentation des apports français dédiés à la venue d'étudiants étrangers dans notre pays. Vous l'avez compris, cet amendement vise à sortir les frais d'écolage du champ de l'aide publique au développement. Michelle Gréaume. Une nouvelle fois, on doit s'interroger sur ce qu'est le coeur de l'aide publique au développement. Si l'accueil des réfugiés est une nécessité, sa comptabilisation en aide publique au développement pose question à plusieurs titres : premièrement, elle gonfle artificiellement l'aide apportée aux populations locales ; deuxièmement, nous devons nous interroger sur la pertinence d'une telle comptabilisation. Il est vrai, monsieur le ministre, que l'idée base de l'OCDE, mais elle reste d'application volontaire. En effet, les règles du Comité d'aide au développement autorisent les pays à comptabiliser en APD certaines dépenses en rapport avec les réfugiés, mais elles n'en font aucunement une obligation. C'est bien la France et, plus largement,

et, d'autre part, à prendre en considération les derniers développements relatifs au nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour 2021-2027, lequel crée un instrument de voisinage, développement et de coopération internationale qui comprend les dépenses de l'Union en matière de développement international.

Comme je l'ai déjà évoqué, les peuples habitant ces territoires sont particulièrement vulnérables face aux projets de protection de la biodiversité, qui reposent sur une conception excluant toute présence et toute activité humaines. De la même manière, ces populations sont exposées à différentes formes d'accaparement des terres,

les mécanismes de conservation fondés sur la gestion communautaire par les peuples autochtones. Cet amendement vise à assurer la cohérence entre les politiques publiques ayant un impact sur les ODD, les objectifs de la politique de développement

et l'assainissement 2020-2030 n'est intégrée dans la priorité sectorielle n° 4 sur l'eau et l'assainissement. À la suite d'une demande du Cicid, la France a adopté cette nouvelle stratégie internationale en stratégie internationale en février 2020, après un processus de consultation d'un an et demi, piloté par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et impliquant de nombreux acteurs. La stratégie constitue un document d'orientation politique pour l'action extérieure de la France dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Cette action poursuit, d'après le document, deux objectifs : l'accès universel et équitable à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, et la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des bassins versants. Cet amendement vise à intégrer cette référence à l'alinéa 93 du rapport annexé.

vise à clarifier nos engagements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, en prévoyant notamment une augmentation de nos dons à ce secteur et en inscrivant une référence à la stratégie internationale de la France pour l'eau et l'assainissement 2020-2030, qui a été adoptée en février 2020. nous semble cohérente dans la mesure où les autres priorités sectorielles identifiées dans le CPG reposent sur les stratégies existantes dans leur secteur, ce qui contribue à les renforcer. La stratégie doit orienter notre action extérieure dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, secteur essentiel de l'aide publique au développement. Ses recommandations sont cohérentes avec les grandes orientations du texte. Le document reconnaît la prépondérance néfaste de l'instrument des prêts : en 2019, 87 % des versements bilatéraux pour ce secteur se faisaient sous cette forme,

et 2019. Cela est tout à fait regrettable, car l'accès à l'eau et aux installations sanitaires est essentiel dans les pays les plus pauvres ou en crise, qui ne peuvent rembourser des prêts. Il faut donc prévoir une meilleure répartition des dons dans ce secteur.

L'assainissement reste un enjeu majeur quand l'on sait que, selon les données de l'OMS et de l'Unicef, 2,4 milliards de personnes n'ont pas d'accès élémentaire à une installation sanitaire et que 1 milliard d'entre elles Or l'accès à ces installations réduit de plus de 30 % la morbidité diarrhéique et impacte fortement la nutrition, l'accès à l'éducation ou l'égalité des genres. Au regard de ces enjeux, pourquoi ne pas faire mention de la stratégie française déjà adoptée en la matière ?

président de la commission. Au terme de cette deuxième partie de débat, je voudrais adresser quelques remerciements. Nous aurons l'occasion à l'issue du débat, lorsque le vote interviendra, d'en tirer les leçons et de montrer comment le Sénat a enrichi ce texte. En attendant, je veux d'ores et déjà remercier la présidence, le ministre pour sa qualité d'écoute et la dimension constructive qu'il a donnée à nos échanges et, surtout, nos collègues, singulièrement celles et ceux qui n'appartiennent pas à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Certes, la matière est assez technique, mais il s'agit tout de même d'une affaire de l'ordre de 15 milliards d'euros. Ce montant n'est pas tout à fait sans importance et participe très largement de l'aide que la France,